L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

et ce notamment quand un risque majeur existe du point de vue de l'intégrité physique du demandeur d'asile. Comme les évolutions du droit y ont conduit, nous avons de fait laissé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, le soin de fixer de manière régulière la liste des pays dits « sûrs », c'est-à-dire ne permettant pas de justifier d'une demande d'asile auprès des services français. La liste des pays sûrs recouvre, selon l'OFPRA,

Or la liste concernée n'a guère évolué dans la dernière période et comprend des pays où tout n'est pourtant pas si simple, notamment dès qu'il s'agit de certaines situations personnelles. personnelles. Des pays sûrs pratiquent en effet la discrimination à l'endroit des homosexuels, sans parler de la place de la femme dans certaines sociétés ... De manière plus générale, la liste des pays sûrs comprend des pays ayant été au centre de la démarche de plusieurs associations de défense des travailleurs étrangers et des demandeurs d'asile. Je vous épargne la situation, d'une extrême gravité, dégradante, humiliante, inhumaine, dans certains pays tels que l'Arménie, l'Albanie, la Géorgie, la Serbie ou le Kosovo, qui justifie à elle seule l'adoption de cet amendement.

D'un point de vue légistique, on connaît les limites des dispositions fonctionnant à partir de listes et les doutes qui planent toujours quant à leur exhaustivité. Sans y déroger, la notion régie par l'article L. 722-1 du code de l'entrée Depuis 2015, le CESEDA prévoit que la liste est revue régulièrement par le conseil d'administration de l'OFPRA. Or la liste des pays sûrs n'a pas été actualisée depuis 2015. L'objet de cet amendement est donc de garantir une révision tous tous les six mois afin de parer à d'éventuels basculements et d'éviter le renvoi précipité de certains demandeurs alors même qu'ils courent un risque chez eux.

de la liste des pays considérés comme d'origine sûrs. L'obligation actuelle de réexamen régulier me semble pourtant satisfaisante, et mieux adaptée aux besoins et à la situation. D'ailleurs, le conseil d'administration peut déjà, en cas d'évolution rapide

réglementaire qui n'est pas tout à fait à la mesure du problème. Au fond, l'ordre international, qui se traduit par beaucoup de désordres et de conflits, fait évoluer jour après jour la situation des pays sûrs. Il est vain d'embouteiller le conseil d'administration de l'OFPRA en lui demandant de réexaminer intégralement la liste des pays sûrs tous les six mois. Ne croyez-vous pas qu'il a mieux à faire en définissant la stratégie de l'OFPRA et en discutant avec le Gouvernement des moyens mis à sa disposition pour assurer la bonne exécution de ses missions ? C'est à tout moment,

de notre pays. Je vous en supplie, concentrons-nous sur l'essentiel, de sorte que nous puissions avancer et que notre débat ait toute la dignité requise pour convaincre les Français, qui le suivent, de la force des propositions du Sénat.

Si nous étions à Berlin hier, c'était à la fois pour faire avancer l'Europe du point de vue économique, puisque

Lorsque l'on examine ce qui a permis au niveau européen de faire baisser les flux migratoires, on s'aperçoit que ce sont d'abord les accords que nous avons su passer avec un certain nombre de pays.

venant soit de la Corne de l'Afrique, d'Érythrée ou d'Éthiopie, soit de l'Afrique occidentale, se retrouvant à Agadez. Un certain nombre de migrants ont fait la traversée du désert,

de 1,2 milliard à 2 milliards d'ici à 2050. Penser que ces 2 milliards de personnes pourraient venir ici est totalement illusoire.

Cet amendement vise à introduire une procédure exceptionnelle de suspension d'un pays de la liste des pays d'origine sûrs, mise en oeuvre exclusivement par le directeur de l'OFPRA, puis confirmée par le conseil d'administration.

de défense des droits des femmes ou de défense des droits des enfants de saisir le conseil d'administration de l'OFPRA d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un État de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Complété en commission des lois par un amendement de nos collègues socialistes, le texte prévoit désormais d'accorder ce droit aux associations de défense des personnes homosexuelles et transgenres. Ces amendements ont fort heureusement été adoptés par la commission des lois, en cohérence avec la protection accordée aux personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Nous estimons cependant que ces avancées ne sont pas satisfaisantes en l'état et souhaitons remplacer la mention « personnes homosexuelles ou transgenres » par « personnes LGBTQI », afin que les bisexuels et les intersexes soient protégés au même titre. Le cas des personnes bisexuelles est particulièrement préoccupant comme nous l'ont confié les associations de défense des personnes LGBTQI que nous avons auditionnées ces dernières semaines. Les bisexuels se voient en effet souvent refuser une demande de séjour au titre des persécutions subies de par leur orientation sexuelle, car ils auraient eu par le passé ou des compagnes du sexe opposé. Le terme « LGBTQI » permettrait d'offrir une protection plus effective et inclusive à ces requérants, qui subissent de nombreuses violences et persécutions dans leur pays d'origine. monsieur le rapporteur,

M. Guillaume Gontard. Sous couvert de simplification administrative, l'article 5 du projet de loi autorise l'OFPRA à adresser la convocation à l'entretien individuel « par tout moyen », y compris électronique : messages téléphoniques, courriels, et j'en passe. Sans entrer dans des considérations juridiques, si j'en appelle d'abord au bon sens, chacun peut entendre que cette mesure est parfaitement injuste et s'inscrit dans une logique purement comptable. Cette liberté dans la transmission des informations se fera inévitablement au détriment des demandeurs d'asile, étant donné leur situation particulièrement vulnérable et leurs conditions de vie précaires,

Aucune disposition ne garantit que la décision ne soit pas opposée lorsqu'il n'est pas certain que le demandeur ait pu en prendre personnellement connaissance. D'ailleurs, comme le souligne dans son rapport François-Noël Buffet, l'OFPRA note qu'il existe actuellement de nombreux dysfonctionnements dans la réception effective des convocations ou des notifications de décision par les demandeurs d'asile. Pensez-vous donc sérieusement que ces nouvelles modalités d'envoi « par tout moyen » amélioreront la situation ? En outre, ce mode d'envoi de la convocation ne respecte pas le principe de confidentialité, que le Conseil constitutionnel a érigé au rang de garantie essentielle du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle impliquant que les demandeurs d'asile bénéficient d'une protection particulière. Le présent amendement prévoit donc d'envoyer systématiquement la convocation et les décisions de l'OFPRA par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par tout moyen, comme le permet le projet de loi. Les dispositions adoptées en commission des lois à l'Assemblée nationale qui encadrent cette autorisation n'apportent pas de garanties suffisantes au regard de la situation particulièrement précaire des demandeurs d'asile. Les précisions souhaitées par la commission des lois du Sénat et renvoyées à un décret en Conseil d'État sont également loin d'être satisfaisantes. Seule la voie postale permet le contrôle de l'envoi et de la bonne réception de la convocation ou des décisions par les intéressés et garantit, donc, l'efficacité de la transmission des informations aux demandeurs d'asile.

garantit non seulement la réception par le demandeur des documents qui lui sont envoyés, en particulier les notifications, mais aussi sa compréhension. Rappelons que plus de la moitié des demandeurs d'asile n'ont pas hébergement ; ils sont domiciliés dans des plateformes d'accueil ou chez des associations, qui ont mis en place des dispositifs pour les alerter lorsqu'ils reçoivent un courrier. Ces plateformes et ces associations insistent sur la nécessité d'accompagner le demandeur afin qu'il comprenne les documents qu'il reçoit, en particulier les notifications, et de lui permettre dès réception, si les délais sont réduits, d'engager les démarches utiles pour répondre à une convocation ou, plus important encore, engager un recours. Si la voie dématérialisée, telle qu'elle est préconisée par l'Assemblée nationale, peut sembler plus simple, il n'en reste pas moins que son efficacité pose problème. Le Conseil d'État a donc, dans son avis, proscrit les envois automatiques. Si l'amendement déposé par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste n'était pas adopté, il conviendrait alors

a considéré que si ces deux éléments n'étaient pas garantis, on pourrait considérer, d'une part, que les notifications sont incertaines et, d'autre part, qu'elles pourraient porter atteinte au caractère équitable de la procédure.

cet amendement vise à laisser à l'Office de plus grandes marges de manoeuvre dans sa décision de clôture des dossiers. Depuis la loi du 29 juillet 2015, l'OFPRA a la possibilité de clôturer des dossiers de demande d'asile dans plusieurs cas, notamment lorsque la personne concernée retire sa demande d'asile, à l'occasion d'un entretien ou par courrier, lorsqu'elle n'a pas introduit sa demande dans le délai de 21 jours, lorsqu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien ou encore lorsqu'elle n'a pu être contactée, faute d'avoir transmis son adresse à l'Office dans un délai raisonnable. En raison des difficultés pratiques déjà évoquées et liées aux mauvaises conditions d'hébergement des demandeurs d'asile, il est probable que ces situations soient fréquentes. Il semble donc que cette disposition produise des effets limités dans une perspective de désengorgement de l'OFPRA, alors même qu'elle pourrait donner lieu à des clôtures de dossiers de demande d'asile légitimes et avoir des conséquences négatives sur l'activité de l'OFPRA, celle des préfectures. En effet, le CESEDA permet aux demandeurs d'asile de solliciter auprès de l'OFPRA la réouverture de leur dossier, dans les neuf mois suivant la décision de clôture. Selon le dernier rapport d'activité de l'Office, ces réouvertures sont peu nombreuses, preuve de l'utilisation pertinente de cette facilité par l'OFPRA. On en comptait 30 en 2016, puis 142 en 2017. II est à craindre que la clôture automatique donne lieu à une augmentation considérable des demandes de réouverture de dossier, ce qui aurait le défaut de toucher non seulement l'OFPRA, mais également les préfectures.

la certitude de la réception par le demandeur. C'est la raison pour laquelle la commission des lois, conservant le dispositif mis en place par le Gouvernement, qui lui paraît utile,

le demandeur n'a pas introduit, sans motif légitime, sa demande d'asile ; la clôture lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions d'accueil et d'hébergement, introduit par la commission- ce cas est conforme à l'article 28 de la directive Procédures et est de nature à dissuader les demandes d'asile abusives demandes d'asile abusives - ; enfin, s'agissant de la compétence liée de l'OFPRA en cas de retrait d'une demande d'asile par un demandeur, il semble logique de prévoir alors la clôture du dossier. En effet, dès lors que les conditions d'application de cet article sont réunies, l'OFPRA doit décider,

suis donc tout à fait sur la ligne de la commission et du Gouvernement : laisser traiter les dossiers par l'OFPRA explication de vote. La réduction des délais était absolument nécessaire, personne ne le conteste. D'ailleurs, elle a commencé bien avant. On a atteint un pic

Les amendements qui sont présentés visent simplement à ne pas restreindre les droits en la matière. Si vous voulez accélérer la procédure en restreignant les droits à tous les étages, vous allez multiplier les situations d'injustice

Il fixe notamment les modalités permettant d'assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » Les choses sont donc parfaitement claires

Elle repose sur l'idée selon laquelle la réduction des délais de la procédure de demande d'asile est plus protectrice pour les personnes concernées. Or, s'agissant de procédures très complexes et de personnes très vulnérables, cet argument peut être remis en cause. Lors des visites que nous avons conduites pour préparer l'examen de ce projet de loi, nous avons pu constater le désarroi des personnes sollicitant une protection internationale face à un système bureaucratique très élaboré et codifié. Dans plusieurs pays d'origine de ces demandeurs d'asile, comme en Afghanistan, la culture administrative est diamétralement opposée à la nôtre, ne serait-ce qu'en matière d'identification des personnes. Certaines questions qui paraissent aussi banales que l'identification par la date de naissance n'ont aucun sens dans certains pays. Si cette réforme, comme les précédentes, porte essentiellement sur la fluidification des procédures devant l'OFPRA et la CNDA, les dispositifs en amont de la saisine de l'OFPRA sont sous-dimensionnés au regard du nombre de demandes d'asile et reposent en grande partie sur le travail associatif de nombreux bénévoles. Dans ces conditions, il paraît nécessaire de laisser une période suffisante à ces personnes pour se préparer à la complexité de la procédure, au risque d'écarter les demandes légitimes et de favoriser les demandes dilatoires déposées par des individus plus familiers du système bureaucratique français. L'amendement n° 39 rectifié,

Ces alinéas 7 à 9 prévoient dix nouveaux cas pour lesquels la procédure accélérée serait prévue dans le traitement des dossiers. Mes chers collègues, vous le savez, la procédure accélérée ouvre des possibilités moindres pour le requérant de monter un dossier lui permettant d'obtenir un titre de séjour. un titre de séjour. Nous estimons que, au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle. La question de l'attribution du droit d'asile ou d'un autre titre de séjour est une question sérieuse qui nécessite un examen minutieux des dossiers déposés à l'OFPRA.

accélérée soit limitée aux seuls cas de fraude sur l'identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut-Commissariat aux réfugiés et aux demandes d'asile en rétention. Cette limitation devrait permettre que la procédure normale ne relève désormais plus du domaine de la justice d'exception.

Alors que les mineurs non accompagnés sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, aucune garantie procédurale particulière n'est prévue dans le traitement de leur demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Ainsi, leur particulière vulnérabilité n'empêche pas le recours à la procédure accélérée, plus courte de six mois par rapport à la procédure dite « normale », pour examiner leur demande d'asile quand ils sont originaires d'un pays considéré comme sûr ou que leur présence en France est considérée comme comme constituant une menace grave pour l'ordre public. À défaut d'une procédure véritablement protectrice de leurs droits, le bénéfice d'une procédure normale est un minimum qui devrait leur être garanti au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel l'article L. 741-4 du CESEDA se réfère pourtant. Pour cette raison, nous demandons que les enfants ne puissent pas faire l'objet d'une procédure accélérée et qu'ils bénéficient de toutes les garanties d'une procédure de droit commun permettant un réel examen de leur situation.

-pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée et sous une fausse identité. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France en considérant que cet élément ne discréditait pas l'ensemble des

de M. Leconte. L'article L. 723-2 du CESEDA prévoit qu'il sera statué en procédure accélérée lorsque le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de 120 jours à compter de son entrée en France.

présenter l'amendement n° 42. Cet amendement vise à préserver la durée actuelle de 120 jours. Le mieux est parfois l'ennemi du bien et vitesse ne doit pas être confondue avec précipitation. C'est évidemment ce qui ressort de l'analyse de l'article 5 quand il s'agit des délais d'instruction des demandes d'accession au statut de réfugié politique, qui ne peuvent, de notre point de vue, souffrir d'approximations. vrai qu'il nous faut respecter la lettre et l'esprit du texte de la convention de Genève. À son article 31, il est précisé s'agissant des réfugiés en situation irrégulière : « Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. « Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable, ainsi que toutes facilités nécessaires. » Un délai raisonnable, nous dit donc la convention, dont notre pays fut, faut-il le rappeler, l'un des initiateurs et qui a servi de base juridique à la création de l'OFPRA. Il faut dire que la reconstitution d'un parcours personnel et d'une existence, même quand on a vingt ans, ou moins, et que l'on vient d'un pays en guerre dépourvu de la moindre once d'administration en état de marche, n'est pas forcément l'exercice le plus simple et le plus commode. Il est pour nous hors de question que, au nom d'un droit d'asile effectif, de sordides considérations comptables ou des impératifs de productivité apparente du travail des fonctionnaires et assimilés de l'OFPRA prennent prennent le pas sur les obligations que notre pays se doit d'accomplir, eu égard à ses engagements internationaux déjà anciens. Opposer des contraintes budgétaires au plein exercice du droit international n'est pas acceptable. Tel est le sens de cet amendement de notre groupe, que nous ne pouvons que vous inviter à adopter. La 201 rectifié. Cet amendement a vocation à supprimer l'abaissement à 90 jours du délai dans lequel un demandeur d'asile doit présenter sa demande, sous peine de la voir examinée en procédure accélérée. Cet abaissement du délai ignore les conditions de détresse dans lesquelles peuvent arriver certains réfugiés et le parcours d'obstacles que constitue le dépôt d'une demande d'asile pour des personnes venant de pays où l'administration est sans doute moins élaborée que celle de notre pays. En trois mois, ces réfugiés devront se mettre à l'abri, se nourrir, recevoir le cas échéant les soins nécessaires et entreprendre les indispensables connaître les guichets auxquels s'adresser- bref, tout ce que nous connaissons, nous, par coeur ! Cet abaissement du délai à 90 jours a pour seul objectif de faire examiner en procédure accélérée un nombre accru de demandes de protection, alors même que 40 % des demandes sont déjà examinées en procédure accélérée. Avec ce texte, plus d'un dossier sur deux sera examiné en procédure accélérée ; moins de la moitié des demandes sera examinée en vertu de la procédure de droit commun.

et appauvrissant davantage nos compatriotes déjà dans la difficulté. Cet amendement vise à réduire le délai à partir duquel l'administration peut recourir à la procédure accélérée d'examen de la demande d'asile. Diminuer celui-ci de 120 à 90 jours n'est évidemment pas suffisant. Qu'un étranger n'ait pas demandé l'asile 20 jours après son arrivée clandestine signifie clairement que la procédure d'asile a été détournée. Aujourd'hui, rien n'oblige un demandeur d'asile entré de façon irrégulière sur le territoire national à déposer sa demande avant un délai de quatre mois, soit 120 jours, et qui, si le projet de loi est adopté, sera demain de 90 jours. Passer de 120 à 90 jours ne réglera pas la situation extrêmement complexe à laquelle nous sommes confrontés. Sur 100 000 demandes d'asile, je le rappelle, 43 000 sont acceptées en moyenne chaque année. Mais tous les déboutés, ou presque, restent sur le territoire national. Nous devons juguler le phénomène migratoire, et cela passe par une véritable exigence en matière de droit d'asile. Dans cette optique, nous pouvons et nous devons réduire les délais à 20 jours. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, madame la présidente. l'article 14 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale

1810 du 15 avril 2011 concernant les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe prévoit de nombreux droits et garanties à leur profit. Parmi eux figurent le respect de l'enfant, la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdiction du refoulement, l'accès aux procédures d'asile, l'interdiction de la rétention d'enfants migrants, la recherche de solutions durables et le regroupement familial. Cette résolution insiste également sur le caractère humanitaire devant prévaloir dans le traitement des enfants migrants non accompagnés. À cet effet, elle dispose que les États doivent porter plus d'attention à la protection des enfants qu'au contrôle de l'immigration. C'est pourquoi cet amendement vise à introduire dans la loi l'interdiction absolue

s'il a présenté une demande de réexamen ou si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. L'intérêt supérieur du mineur exige un examen bénéficiant de toutes les garanties procédurales, ce qui n'est pas le cas dans la procédure accélérée

Cet amendement a vocation à revenir sur une disposition insérée par la commission des lois. Aujourd'hui, l'OFPRA, dont on ne cesse de louer la compétence, l'efficacité, l'intelligence, a la possibilité de statuer en procédure accélérée dans un certain nombre de cas. L'amendement vise à supprimer cette obligation lorsque la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.

Il se peut, en revanche, dans le cadre d'une décision judiciaire, celle du juge des enfants, qu'ils soient obligés de retourner dans leur pays d'origine s'ils peuvent y être accueillis par leur famille ou un tuteur légal. Dans ces conditions, les droits du mineur sont parfaitement assurés. Les choses sont claires pour la commission, qui a

L'amendement n° 206 rectifié tend à prévoir que l'absence d'entretien pour raisons médicales n'influe pas dans un sens défavorable la décision de l'OFPRA. que l'OFPRA applique effectivement cette disposition et adopte des dispositions réglementaires en interne, il ne semble pas opportun de faire figurer cette précision dans le texte,

202 rectifié vise à supprimer l'obligation faite à l'OFPRA, introduite en commission, de statuer en procédure accélérée, lorsque la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Il semble parfaitement logique, à partir du moment où l'autorité administrative

qui prévoit, en particulier, que les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, de traiter en procédure

postdatée ». J'attendais de votre part une vision générale, qui permette d'introduire un peu de rationalité dans notre débat. Malheureusement, vous en êtes resté à une analyse éminemment comptable, technique, évoquant la manière dont il faut gérer les autorisations.

en rappelant plusieurs points fondamentaux. Premièrement, les flux migratoires n'ont jamais été aussi peu importants en France. Deuxièmement, la présence des immigrés en France n'a jamais été aussi faible- c'est l'une des plus faibles des pays de l'OCDE. Troisièmement, les immigrés ne viennent pas des pays les plus pauvres. Quatrièmement, les immigrés qui arrivent en France ne sont pas les plus pauvres : au contraire, ils ont très souvent un niveau de formation élevé.

observé en 2017 montre à l'envi que nous ne disposons pas des moyens matériels et humains d'instruire correctement ces dossiers. À notre avis, cette situation trouve son origine dans deux faits essentiels : d'une part, une insuffisance des moyens pour traiter convenablement les demandes d'autre part, l'information sans doute parcellaire dédiée aux hommes et aux femmes qui candidatent au statut de réfugié, ne leur assurant pas la pleine maîtrise de leurs droits. On retrouve, à l'article 5, ce que le Défenseur des droits a, à juste titre, dénoncé dans ce texte, à savoir le climat de suspicion généralisée, opposé par principe à toute demande d'asile, faisant fi des parcours personnels d'individus souvent aux prises avec des contraintes géopolitiques qui les dépassent.

Si je puis me permettre cette comparaison, on en sait quelque chose au Parlement. Votre texte permettra que les demandes soient examinées en un temps record. Nous considérons, à l'instar de la majorité des associations

est ainsi libellé : La parole est à Mme Maryse Carrère. Le projet de loi donne la possibilité à l'OFPRA d'adresser au demandeur d'asile la convocation à l'entretien individuel et de notifier ses décisions écrites « par tout moyen », ouvrant ainsi la possibilité d'un envoi par voie dématérialisée. répond à une préoccupation de l'OFPRA, qui éprouve souvent des difficultés pour adresser ses convocations. Dans le droit administratif français, la notification est pourtant un élément procédural essentiel. Dans son avis du 15 février 2018, le Conseil d'État, se prononçant sur le présent projet de loi, a ainsi alerté le législateur sur les risques liés à une notification « par tout moyen » : « Le plus grand soin devra toutefois être apporté au choix des moyens techniques de sorte qu'une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que dans la mesure où il est démontré qu'elle a été opérée personnellement et qu'il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l'intéressé. À défaut, la combinaison d'un délai très bref avec des modalités incertaines de notification pourrait être regardée comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure. Or, comme certains de nos concitoyens, les demandeurs d'asile sont eux aussi confrontés à la fracture numérique. Qu'ils soient hébergés ou non, la grande majorité d'entre eux n'ont pas un accès facile à internet. La plupart des centres d'hébergement ne sont pas suffisamment équipés, faute de moyens.

met ainsi en oeuvre une disposition de la directive Procédures, que nous avons déjà évoquée, laquelle prévoit que, lorsqu'aucun entretien personnel n'est mené pour raisons médicales, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à son représentant de fournir davantage d'informations. Cet amendement a été rectifié, notamment pour encadrer cette nouvelle garantie dans le temps et pour prévoir que l'Office, lorsqu'il décide de se dispenser d'entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé, informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu'il jugerait utile.

aux demandeurs dont les facultés de compréhension et d'expression écrites ne sont pas altérées un questionnaire écrit personnalisé afin de recueillir les éléments complémentaires utiles

Il s'agit, en effet, du premier obstacle pour le demandeur d'asile, lequel place une partie de son sort entre les mains des interprètes qui lui sont assignés le jour de son entretien, puis lors de son audience. Le présent projet de loi prévoit de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d'asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure. Il s'agit d'une restriction à l'exercice du droit du demandeur d'asile à être entendu dans une langue qu'il comprend. En effet, un demandeur d'asile peut être amené à déclarer qu'il comprend une langue sans la maîtriser entièrement. Or exposer son histoire, surtout si elle est douloureuse et compliquée, et comprendre les subtilités de questions posées au cours d'un entretien en vue d'examiner un besoin de protection supposent une maîtrise linguistique qui va bien au-delà de la simple compréhension de phrases courtes de la conversation courante. Une erreur dans la déclaration aurait aussi d'importantes conséquences pendant toute la durée de la procédure. Quel est l'avis de la commission ?

est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à modifier la définition de la langue de la procédure de demande d'asile, telle qu'elle est aujourd'hui mentionnée à l'article L. 723-6 du relatif à l'entretien personnel. La directive Procédures prévoit, dans son article 15, que la communication, lors de l'entretien personnel, doit avoir lieu « dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend ou dans laquelle il est à même de communiquer clairement ». Ces dispositions ont été transposées, en 2015, à l'article L. 723-6 du CESEDA, relatif relatif aux conditions de l'entretien personnel, qui dispose que le demandeur « est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». Le texte ne modifie pas ces termes, qui sont tout à fait conformes à la directive Procédures.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à garantir que le demandeur d'asile sera entendu, au moment de son entretien devant l'officier de protection de l'OFPRA, dans la langue dans laquelle il peut se faire comprendre. Cet entretien est sans doute l'étape la plus essentielle pour le demandeur d'asile, celle au cours de laquelle il fera le récit de son histoire, de ses persécutions et de son parcours. Cela exige d'assurer que le demandeur pourra utiliser une langue qui lui permet de se faire comprendre, c'est-à-dire de pouvoir utiliser un vocabulaire suffisamment précis et subtil. Dès lors, il n'est pas acceptable que l'entretien puisse se faire, comme le prévoit le projet de loi, dans une langue dont le demandeur d'asile a une connaissance « suffisante Avoir une connaissance suffisante ne signifie pas nécessairement être en mesure de se faire correctement comprendre par l'autre. Nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à avoir une connaissance suffisante de l'anglais,

Le scrutin est ouvert.

L'asile interne permet de rejeter une demande d'asile lorsque la personne concernée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine. Les dispositions de cet amendement indiquent que la protection accordée dans le pays doit être non temporaire.

se faire oralement lors de l'entretien ou à tout moment par écrit.

devra être considérée, non comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile pleine et entière. En raison des changements qui ont pu se produire dans cet intervalle de trois ans, tant pour le demandeur que dans le pays dont il est originaire, il nous paraît nécessaire de garantir au demandeur que sa demande bénéficiera de toutes les garanties liées à un examen de droit commun et non d'un examen qui pourrait être considéré comme étant « au rabais Monsieur le rapporteur,

en prévoyant qu'est considérée ainsi toute nouvelle demande présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Cette procédure a été conçue pour traiter le plus rapidement possible des demandes pouvant apparaître comme manifestement dilatoires, tout en assurant la garantie des droits des demandeurs qui apporteraient des faits nouveaux à la connaissance de l'OFPRA. L'Office va ainsi apprécier la nouveauté et la portée des arguments invoqués par le demandeur afin de déterminer s'ils

ce dont nous avons eu parfois l'occasion de nous réjouir.

les discriminations en raison de l'orientation sexuelle et de l'origine ethnique, les violences faites aux femmes et aux mineurs, notamment la traite de personnes, les entraves au droit d'asile, les entraves à la liberté d'expression, les pratiques de vendetta. En Géorgie persistent les traitements inhumains et dégradants, la détention arbitraire. La situation des minorités sexuelles, ethniques et religieuses y est notamment problématique. En Serbie règne encore une corruption endémique, de sorte que l'État de droit n'y est pas garanti. Les traitements inhumains de la part de la police sont fréquents. La situation des minorités ethniques, notamment des Roms, est préoccupante. Les discriminations en raison de la religion, du handicap ou de l'orientation sexuelle, ainsi que les violences faites aux femmes et aux mineurs, sont monnaie courante. Le droit d'asile y est méconnu. Au Kosovo, la corruption et la criminalité organisée règnent. Le fonctionnement des institutions de l'État de droit, à commencer par la justice, est défaillant. Les discriminations en raison de l'orientation sexuelle et les violences à l'égard des homosexuels sont préoccupantes. Les minorités ethniques sont dans une situation déplorable. La liberté de la presse n'est pas garantie, et les journalistes font l'objet de menaces. Les femmes et les mineurs sont victimes de violences spécifiques. Le Kosovo est à la fois une source et une destination du trafic d'êtres humains.

compte tenu des évolutions que connaissent les pays du sud-est de l'Europe, il est effectivement souhaitable que l'Union européenne continue

La composition actuelle du conseil d'administration de l'OFPRA, telle que prévue par l'article L. 722-1 du CESEDA, favorise très largement la représentation de l'État, ce qui peut constituer un problème à nos yeux. Ainsi, le conseil d'administration comprend aujourd'hui deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget, soit, au total, dix représentants de l'État. Même le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du ministre chargé de l'asile. Siègent également deux membres du Parlement européen, ainsi qu'un représentant du personnel de l'OFPRA, élu pour trois ans par les agents de l'Office,

attribuées à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, nous souhaitons que le président de celle-ci prenne part aux délibérations du conseil d'administration de l'OFPRA, avec voix consultative. L'amendement

en s'inspirant de la proposition n° 2 du rapport d'information sur la procédure de demande d'asile remis en novembre 2012 par MM. Jean-Yves Leconte et Christophe-André Frassa.

Gouvernement ? Le Gouvernement n'est pas favorable à ce que l'on change la composition du conseil d'administration de l'OFPRA,

dans leur pays en raison de leur action en faveur des droits des femmes, de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. Notre groupe a récemment été sollicité par une femme dénoncée par son mari pour avoir organisé une exposition artistique d'oeuvres jugées illégales. son pays lui vaudrait une peine d'emprisonnement. Bien que les femmes puissent être persécutées dans leur pays pour les mêmes raisons que les hommes, la forme de ces persécutions revêt un caractère particulier, lié à leur genre. Les contraintes sociales pèsent plus fortement sur les femmes et les exposent à de nombreuses violences. Je veux y insister. Toute action est un combat. Elles sont emprisonnées pour s'être mêlées de la vie politique, assassinées pour avoir refusé un mariage, violées parce que non hétérosexuelles ou tuées pour avoir lutté en faveur de l'égalité. Les femmes représentent la moitié des 244 millions de migrants dans le monde. À la dangerosité du voyage s'ajoute l'incertitude à l'arrivée dans le pays d'accueil, où elles se trouvent une fois encore particulièrement exposées. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes du 18 décembre 2017 a souligné les nombreuses difficultés auxquelles les femmes demandeuses d'asile doivent faire face. Notons qu'elles ne représentent que 33 % des demandeurs d'asile. La loi doit considérer que toutes les violences qu'elles subissent concernent les politiques publiques et ne sont pas du ressort de la vie privée. Alors que de plus en plus de femmes osent s'exprimer, dans leur pays, pour l'égalité des droits et contre les violences dont elles sont la cible,

Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre Mme Cohen. Le statut de demandeur d'asile protège les victimes de persécutions,

que les droits des femmes sont respectés et promus dans notre pays et que celles et ceux qui luttent pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les persécutions liées

vise à reconnaître la qualité de réfugié aux femmes persécutées en raison de leur action en faveur des droits des femmes. L'intention est bien sûr sûr louable, mais cette demande me semble satisfaite par le droit en vigueur au titre de l'asile conventionnel défini par la convention de Genève, qui permet d'octroyer l'asile « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA renvoient à cet article de la convention de Genève ainsi qu'à la directive Qualification, qui précise précise les motifs de persécution. L'action en faveur du droit des femmes peut être reconnue comme une opinion politique au sens de la convention de Genève ; la persécution des femmes en tant qu'appartenant à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle est également déjà prise en compte par ladite convention. L'article 10 de la directive Qualification précise d'ailleurs qu' « un groupe social spécifique peut être un

Monsieur le ministre

lois. Mme Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, le sait bien, nous ne nous exprimons pas ici en fonction de notre genre, de nos origines, de nos croyances, de nos professions antérieures.

dans le monde, des pratiques abominables. Je ne sache pas qu'un seul de nos collègues ne soit pas prêt à les dénoncer et à agir pour leur éradication ! Ce n'est pas le sujet. Des actions libératrices courageuses sont menées dans des pays autoritaires qui refusent de reconnaître l'égalité entre les femmes et les hommes et où sont pratiquées un certain nombre d'agressions, comme l'excision, qui sont tout simplement inacceptables.

où l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile auraient décidé de refuser le statut de réfugié à une femme menacée d'excision, à une militante combattant, dans son pays, pour les droits des femmes

Bien entendu, monsieur le président de la commission des lois, j'imagine que tous nos collègues sont prêts à se mobiliser contre l'excision et contre toutes les pratiques cruelles et inhumaines subies par les femmes aux quatre coins de la planète. Mais il n'y a pas que l'excision

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande Le scrutin est ouvert.

2013, la Cour de justice de l'Union européenne établit que les personnes homosexuelles peuvent constituer un groupe social menacé au sens de la convention de Genève sur les réfugiés. Les autorités françaises évaluent le caractère fondé ou infondé de la demande sur la base du récit biographique communiqué à l'OFPRA, de l'entretien conduit par l'officier de protection chargé du dossier et, le cas échéant, du recours soumis à la CNDA. Compte tenu du caractère hautement personnel et intime de ces discriminations, le recours à l'expertise des associations spécialisées est susceptible d'aider les officiers de protection dans l'évaluation des demandes d'asile. Quel est l'avis de la

La commission des lois souhaite que l'OFPRA conserve toute sa liberté et son autorité en matière d'instruction des dossiers, qui sont individuels.

Monsieur le ministre

est à Mme Esther Benbassa. Les causes qui poussent les exilés à s'arracher à leur terre de naissance sont multiples multiples : guerre, instabilité sociale et politique, catastrophe naturelle, discrimination fondée sur le genre ou l'orientation sexuelle, précarité économique

oublier le trajet parcouru par ces exilés. L'évaluation des dossiers se fait sur la base de la situation dans le pays d'origine et du comportement adopté sur le territoire français.

On ne prend conscience de l'ampleur de la difficulté du parcours migratoire que lorsqu'on l'a vécue. Ce n'est probablement le cas que de très peu

C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent d'introduire dans le texte un article prévoyant d'ouvrir le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes ayant subi la torture ou des peines et traitements inhumains

démarches. La fraude à l'asile est très tentante, dans la mesure où les étrangers concernés sont déjà présents sur le territoire français. Il est d'ailleurs très difficile de réunir toutes les conditions pour les reconduire à la frontière. Les chiffres sont accablants

Tous les pays du monde appliquent strictement cette procédure pour les demandes de visa. Nos postes diplomatiques à l'étranger disposent de services suffisamment étoffés pour traiter les demandes de visa d'entrée en France ; il suffira de les mandater pour traiter les demandes d'asile. Nous ne voulons plus de procédures trop longues et coûteuses pour retrouver ceux qui, déboutés du droit d'asile, ont disparu dans la nature- sans

tous ces déboutés ont un toit au-dessus de leur tête, tous sont soignés et tous bénéficient des largesses de notre système social, ... N'importe quoi ! ... tandis que 9 millions de nos compatriotes, dont beaucoup sont d'origine étrangère et essayent

De nombreux demandeurs d'asile risquent de renoncer à former un recours contre les décisions de l'OFPRA, et l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle n'apporte aucune garantie, dans la mesure où les avocats désignés disposeront en fait du même temps pour rédiger la requête et introduire le recours, à savoir quinze jours. Par ailleurs, je crains que la réduction du délai, telle qu'elle est proposée, n'entraîne une augmentation du stock de recours en attente d'être jugés- il s'établit aujourd'hui à 25 000, ce qui est

il est assez normal qu'une partie de nos concitoyens adhèrent au repli sur soi. Nous l'avons dit, la solution est européenne. Alors que l'Europe est en crise, que les pays européens se déchirent, que l'Union européenne se délite, la France, plutôt que de promouvoir la solidarité, de la construire, fait comme d'autres pays et se replie sur elle-même. Elle fait

un recours devant la CNDA, c'est la possibilité, pour des personnes certes déboutées par l'OFPRA, mais toujours présumées réfugiées,

Monsieur le ministre d'État, vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez que tout le Sénat vous entende, quelle que soit l'appartenance politique des uns et des autres.

chacun connaît la grande ouverture d'esprit, et M. le rapporteur de la commission des lois, François-Noël Buffet,

d'asile. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison : si l'on ne parvient pas à traiter les dossiers dans des délais assez brefs, que ce soit devant l'OFPRA ou devant la CNDA, nous aurons toujours davantage de demandeurs, et l'opinion

votre proposition, c'est qu'elle constitue un compromis qui ne nous paraît pas efficace. Nous pensons que l'apport de l'Assemblée nationale sur ce point, qui consiste à

qu'un mémoire complémentaire est annoncé dans la requête sommaire, d'inscrire au rôle pour le jugement la demande faite par un débouté du droit d'asile. Nous sommes en train de discuter d'une d'une proposition pétrie des meilleures intentions pour assurer l'efficacité de la gestion de la demande d'asile, mais qui est en réalité assez peu efficace au regard de ce critère, alors

qui ont droit à la protection soient, en l'espace de six mois, intégrés sur notre territoire et que soient déboutés ceux qui n'y ont pas droit.

et n'interdit pas de compléter les motivations en fait et en droit du recours, comme de produire des pièces nouvelles, après son expiration et jusqu'à clôture de l'instruction peut être regardé

la mise en place d'une assistance juridique sur les plateformes d'accueil, qui existe dans de nombreux autres pays européens et mérite de faire l'objet d'une réflexion. Si la condition

au détriment des droits des demandeurs d'asile et des garanties procédurales qui leur sont dues. Ainsi, il est ici porté atteinte, en particulier, au droit de recours effectif consacré par plusieurs normes supralégislatives, notamment rappelées par la directive Procédures concernant l'asile, disposant que « la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins le droit à un recours effectif devant une juridiction ». L'article 46 de cette directive ne fixe pas de délai, mais précise que « les États membres doivent prévoir des délais raisonnables pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif » et que ces délais ne doivent pas rendre le recours « impossible ou excessivement difficile ». Or, en l'occurrence, alors que la commission des lois du Sénat est revenue au droit existant, déjà insuffisant, qui fixe le délai de recours à un mois,

que pour n'importe quel autre justiciable en France ! Cet amendement répond l'objectif fixé par le rapporteur de la commission des lois. Nous l'invitons donc à poursuivre son bon raisonnement en l'adoptant

puisque j'ai proposé à la commission de conserver le délai d'un mois pour interjeter appel d'une décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. Bravo ! Pourquoi l'ai-je fait ?

ceux qui utilisent la procédure de demande d'asile à d'autres fins que celle d'obtenir réellement la protection de ceux qu'ils prétendent protéger. Des efforts ont été faits depuis plusieurs années.

comme en Autriche, en Pologne, en Hongrie ou aux États-Unis, où l'on peut séparer des enfants de leurs parents et les mettre dans des cages

propos de M. le ministre de l'intérieur selon lesquels accueillir trop de demandeurs d'asile, ce serait s'exposer à une menace d'extrémisation des esprits. Ainsi donc, pour éviter l'élection de candidates et de candidats

toute ma considération et tout mon respect pour la tâche essentielle qui est la vôtre et pour votre personne. Après Après avoir rappelé ces fondamentaux qui facilitent notre dialogue, je dois vous dire que vous auriez été, me semble-t-il, plus convaincant si vous n'aviez pas concédé à votre majorité à l'Assemblée nationale

puis le mémoire complémentaire, vous avez réduit à néant votre proposition de ramener à quinze jours le délai d'introduction de la requête. Dans ces conditions, je crois que le plus sage,